monsieur le président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

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (projet n° 567, texte

l'a très justement rappelé hier soir. Dans de nombreux domaines, comme l'aménagement, le tourisme, le développement économique ou la revitalisation des centres-villes, la société publique locale est devenue l'instrument privilégié de la mutualisation et de la modernisation entre collectivités locales de toutes tailles et de tous niveaux, en permettant de concilier 100 % de maîtrise publique et 100 % de d'entreprise. Dans la mesure où les sociétés publiques locales ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, à intervenir dans le champ des missions d'intérêt général, plus particulièrement en matière de logement, il convient d'ajuster les règles de droit existant, afin que les sociétés publiques locales puissent pleinement intervenir dans le domaine du logement social.

Les cotisations que les organismes d'HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, servent, en partie, à alimenter le Fonds national des aides à la pierre, qui contribue au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux, mais qui n'intervient que sur le seul territoire de la France hexagonale.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l'année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité, Le taux applicable s'élève, au maximum, à 2,5 % sur les loyers et à 100 % sur le supplément de loyer de solidarité. Il est proposé ici de supprimer le supplément de loyer de l'assiette

puissiez travailler avec nos collègues d'outre-mer à une meilleure adaptation de leur contribution à la CGLLS. La parole est à M.

Vous avez rendu un arbitrage qui nous était déjà favorable, puisque vous avez refusé l'extension du RLS dans les outre-mer. Pour autant, il ne s'agit pas encore de la bonne solution. Je pense que nous devrions y revenir lors de

L'enjeu des mixités sociales et fonctionnelles est au coeur du projet de loi ÉLAN. Ce texte vise, par ailleurs, à diversifier les sources de revenus des bailleurs sociaux, ainsi qu'à faciliter la production de logements sociaux. Afin de poursuivre cette logique et de pouvoir lutter à la fois contre les ségrégations spatiales et l'habitat insalubre, tout en accélérant les délais de production de logements sociaux, il est nécessaire que les sociétés d'économie mixte participent au processus et puissent le faire en utilisant le mécanisme de la

En fait, ces offices sont des établissements publics locaux. Les dispositions qui les régissent relèvent essentiellement du code de la construction et de l'habitation.

aux acteurs locaux, cet amendement vise à faciliter les recompositions en sécurisant les éventuelles futures opérations de scission des offices. La rédaction proposée s'inspire tout simplement du droit des entreprises et de l'exemple récent de la scission de l'office départemental du Rhône, à la suite de la création de la métropole de Lyon.

comme en droit des sociétés, les créanciers ne peuvent s'opposer à la scission et l'ensemble des droits et obligations attachés à l'ancien office sera maintenu de manière continue dans les nouveaux organismes pour garantir les droits de chacun.

du patrimoine ne relevant pas du logement locatif conventionné à la valeur nette comptable porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des actionnaires, tant publics que privés, ainsi qu'à leur liberté d'entreprendre. Une même valorisation pour l'ensemble du patrimoine ne permet de de garantir ces principes. Le patrimoine ne relevant pas du domaine locatif conventionné doit donc être évalué selon les règles du code de commerce afin de prendre en compte la valeur réelle des activités hors agrément.

dès lors que cela ne remet pas en cause l'objet social de ces derniers. La condition pour permettre ces fusions est que l'évaluation de l'actif soit réalisée dans les mêmes conditions qu'entre les autres organismes, avec des capitaux propres. La règle de valorisation ne s'applique

Cette situation semble aujourd'hui stabilisée, dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs paraissent faire l'objet d'un relatif consensus.

ayant une incidence sur les loyers ou sur les charges locatives, de construction ou de démolition. Nous proposons d'améliorer ce dispositif en ajoutant un alinéa prévoyant une obligation de concertation avec les locataires en cas de regroupement ou de fusion de plusieurs bailleurs. Il s'agit notamment de renforcer l'information sur les décisions pouvant avoir une incidence sur le quotidien des locataires, qui ne doivent pas pâtir des décisions prises par leur bailleur. Ils ne doivent pas se sentir exclus de toute prise de décision les concernant au premier chef. chef. Bien au contraire, leur association par la concertation, ne serait-ce que par leur meilleure information, ne peut être que positive et conduire à des échanges apaisants.

ayant pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts en titres émis par des organismes d'HLM ou conformes au caractère social et territorial du secteur HLM et à l'intérêt économique. Ces fonds pourraient être créés et gérés

ainsi qu'à des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, qui seraient créés à l'initiative de ces groupes ou des offices et gérés directement par eux ou, le cas échéant par l'intermédiaire de sociétés de gestion de portefeuille, partiellement détenues par elles. Tel est l'objet de cet amendement.

investisseurs et l'effort consenti par les finances publiques. Elle a ainsi observé que d'autres dépenses publiques permettaient, à volume égal, d'augmenter plus durablement le parc de logements locatifs. d'illustration, la Cour a calculé que le coût annuel pour les finances publiques d'un logement de 190 000 euros bénéficiant de l'avantage Pinel était, toutes choses égales par ailleurs, trois fois plus élevé que celui d'un logement social comparable, financé par un prêt locatif social, ou deux fois plus élevé que celui d'un logement financé par un prêt locatif aidé d'intégration, alors même que la durée des locations, dans ces derniers cas, est bien supérieure- environ quarante Pour corriger les risques de surproduction en zone détendue, ces aides fiscales ont été progressivement limitées à certains secteurs. Cela a certes permis de concentrer la production de logements aidés sur des zones plus tendues, mais pas nécessairement sur celles où la tension entre l'offre et la demande de logements est la plus forte. Il apparaît même que ces dispositifs rencontrent leur plus forte limite dans ces zones très tendues, où l'accès au logement locatif des classes moyennes est le plus difficile. Ces observations sont directement tirées de l'intéressant rapport de la Cour des comptes sur les aides publiques au logement présentant la forme d'incitations fiscales. La Cour y a notamment relevé la véritable « addiction » des banques et des investisseurs à ces dispositifs d'incitation fiscale. Aujourd'hui, on vend des dispositifs fiscaux par tous les moyens possibles, y compris le canal numérique et cybernétique. On ne propose même plus de logements ... La Cour des comptes produit d'ailleurs, à l'appui de son enquête, deux recommandations d'une part, assurer la mise en déclin des dispositifs existants dont le coût de 1,7 milliard d'euros est à comparer aux 60 millions d'euros du chapitre budgétaire de l'aide à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux

justes et équitables. En effet, les premières études en témoignent, ce n'est pas dans les zones les plus tendues que son efficacité

universelle de patrimoine par voie de fusion, les déficits fiscaux d'une société absorbée sont transférés à la société absorbante à la condition de l'obtention d'un agrément, tel que prévu par l'article 209 du code général des impôts. Or le dernier alinéa du paragraphe de cet article exclut le bénéfice de cet agrément aux sociétés ayant

à la suite notamment des propos de M. Ferrand qualifiant de « faits divers » les actions délictueuses de M. Benalla, adjoint au chef de cabinet du Président de la République. Depuis ce matin, la presse nous livre, heure après heure, des informations nous conduisant à penser que les déclarations du ministre de l'intérieur, hier, devant la Haute Assemblée, étaient à tout le moins bien incomplètes. Vous nous permettrez, monsieur le ministre, d'en être troublés. Pour la sérénité des débats, et afin de restaurer une confiance ébranlée, il nous semble urgent que le ministre de l'intérieur revienne devant notre assemblée, pour nous apporter les compléments d'information que nous sommes en droit d'exiger de lui.

sujet est légitimement posé, et il est normal que le Gouvernement y réponde dans les formes normales du débat démocratique. Pour le reste, sur le dossier lui-même, ayant partagé avec vous ces dernières heures, pour

de la déclaration de M. Retailleau, que nous avons d'ailleurs entendu ce matin sur les ondes, j'ajoute que la commission d'enquête parlementaire ne saurait se réduire à l'audition

ont demandé pourquoi le chef de l'État n'avait pas appliqué, en l'espèce, le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale,

Ils portent une atteinte sévère à la jambe publique du logement social, en favorisant uniquement sa jambe privée. Ils rompent ainsi un modèle spécifiquement français, et mettant en danger les valeurs de la République.

Non seulement il leur est assigné un objectif qui ne correspond pas à leur corps de métier et à leur raison d'être, mais, surtout, ils ne disposeront d'aucun moyen supplémentaire pour mener la tâche qui leur avait été confiée Nous glissons là vers une marchandisation du logement social, puisque les organismes d'HLM sont incités à trouver les moyens de se financer eux-mêmes, dans un contexte déjà très difficile pour eux avec la baisse des APL. C'est donc par la vente de logements sociaux qu'il leur faudra se financer. Nous allons donc vendre notre patrimoine. Les logements les plus anciens seront cédés et deviendront vite des copropriétés dégradées. Les promoteurs, quant à eux, pourront acquérir, dans les quartiers les plus attractifs, des lots qu'ils revendront ou loueront à prix d'or. Ces quartiers deviendront alors rapidement inaccessibles pour beaucoup de nos concitoyens, et la mixité sociale deviendra de fait inexistante. Ainsi, c'est une autre forme d'élitisme et d'entre soi qui est encouragée par ces articles. Encore une fois, l'intérêt privé prime sur l'intérêt général.

d'HLM. Depuis la loi Boutin, la vente du patrimoine a été définie comme un objectif prioritaire pour les organismes d'HLM, objectif largement renforcé par ce projet de loi, puisqu'il est fixé à 40 000 Alors que le pays compte 1,8 million de demandes insatisfaites concernant l'accès à un logement social, nous ne comprenons pas que la vente du patrimoine, donc la perte de logements sociaux, constitue un objectif prioritaire pour ce gouvernement. Au contraire, nous prônons la sanctuarisation de ce patrimoine, au sein d'une agence foncière. Ainsi, à nos yeux, l'objectif prioritaire devrait être d'apporter une réponse aux besoins de construction de logements en zone tendue et de réhabilitation d'un parc parfois dégradé en zone détendue.

d'autres. Parce que les maires disposent d'obligations légales de construction, leur avis doit être conforme, y compris lorsqu'il s'agit de territoires métropolitains. Ainsi, il ne devrait y avoir de ventes de logements sociaux sur un territoire qu'avec l'accord de la commune concernée. On ne peut pas demander aux maires d'atteindre des objectifs de construction et les priver des outils nécessaires pour conserver sur leur territoire un patrimoine locatif social d'ailleurs également d'interdire la vente du patrimoine social dans les communes carencées. Reste que cet article élargit encore inutilement les missions des organismes d'HLM, qui doivent se recentrer sur leur coeur de métier. Il fixe en effet comme un objectif

cela devient la méthode privilégiée et quasiment unique pour financer la construction de parcs nouveaux dans le monde HLM.

auxquelles ne s'appliqueront pas un certain nombre de règles très importantes pour la construction publique,

de 1985. Tout cela va dans le même sens. On nous dit qu'il faut aller plus vite. Pour ma part, j'ai toujours regretté que l'on ne trouve pas des méthodes plus rapides pour mettre en oeuvre les marchés publics, tout en respectant les principes de la concurrence et de l'allotissement. Au bénéfice de cette volonté de rapidité et d'apparente efficacité, on met à mal, d'une part, la qualité, d'autre part, le libre accès à la commande publique et le pluralisme en matière de création architecturale. C'est très grave,

Mme Michelle Gréaume, sur l'article. Cet article 28 du projet de loi est, à n'en pas douter, l'un des pivots du texte, puisqu'il porte sur la définition et les contours des organismes d'HLM. une définition et une nomenclature du secteur locatif social, au sein duquel nous avons vu apparaître une nouvelle catégorie d'opérateurs, à savoir les sociétés de vente de logements sociaux, chargées de ramener dans les caisses les liquidités dont elles ont besoin.

Or la ligne du Gouvernement consiste depuis fort longtemps à favoriser l'aide à la personne, correctif de plus en plus coûteux des désordres du marché, au détriment de l'aide à la construction. On réduit le nombre des organismes d'HLM en escomptant que les économies d'échelle, la restructuration des patrimoines et celle de la dette de chaque organisme ainsi reconstitué suffisent pour permettre à chaque structure de disposer des moyens de son développement. il suffit de lire les attendus et les conditions de mise en oeuvre de la loi de programmation pour observer la faiblesse des crédits destinés à la construction neuve- 50 millions d'euros sont d'euros de moins que le produit de la taxe sur les logements vacants, qui est reversé au budget général -, ainsi que le poids déterminant des aides personnelles, qui sont soumises aux arbitrages budgétaires, et de la dépense fiscale, qui s'élève peu ou prou à 15 milliards d'euros, hors report des déficits fonciers. Les gouvernements, sous M. Sarkozy, avaient beaucoup de défauts ; mais au moins, ils consacraient près de 930 millions d'euros à la construction de logements neufs et à la réhabilitation de logements plus anciens. La captation des ressources du célèbre 1 % patronal, qui est notamment utilisé par l'État pour tenir ses objectifs en termes de rénovation urbaine, ne simplifie guère plus la vie des organismes d'HLM. Tout se passe comme si l'on avait oublié que c'est le mouvement HLM, appuyé par l'épargne populaire collectée au travers du livret A, qui a permis à notre pays de sortir de la crise du logement

leurs activités principales- la construction, l'acquisition, l'amélioration, la gestion et la cession de logements locatifs à loyer modéré -sont déjà exonérées d'impôt sur les sociétés. L'extension des activités exercées par ces organismes à des domaines du logement social qui ne relèvent pas du service public d'intérêt général représente un manquement au principe d'étanchéité des aides publiques et une concurrence déloyale vis-à-vis du secteur privé, qui exerce habituellement ces activités. Selon l'expression de Léon Duguit, est considérée comme relevant du service public « l'activité que les gouvernants doivent obligatoirement exercer dans l'intérêt des gouvernés Les nouvelles activités prévues à l'article 28 ne répondent pas à un tel besoin. Laissons au secteur privé les activités qui lui reviennent ; n'affaiblissons pas l'État en diluant ses ressources dans une concurrence avec ledit secteur privé. La parole

convaincu de la nécessité d'accélérer les processus en matière de passations de marché ; vous nous le répétiez souvent lorsque j'avais l'honneur et le privilège d'être un membre de la commission des lois, que vous présidiez avec la sagacité

engagée il y a de nombreuses années. Et je rappelle que l'objectif auquel nous souhaitons parvenir est de 40 000 logements par an, c'est-à-dire 1 % du parc.

Vous avez osé, monsieur le ministre : ce sont les mots qui nous viennent à l'esprit à la lecture de cet article 28, et singulièrement de la nouvelle définition qu'il donne du secteur HLM, en faisant de la vente de logements locatifs sociaux, dont on est loin de constater qu'ils constituent l'essentiel du parc locatif de ce pays, une activité quasiment ordinaire. Il est vrai que votre gouvernement consacre 60 millions d'euros l'aide à la pierre et 1,7 milliard d'euros à aider les investisseurs immobiliers à optimiser leurs placements financiers aux fins de défiscalisation ! Il n'aura sans doute échappé à personne, ici, que, si l'un des problèmes du marché du travail, en France, réside dans le décalage entre la médiocre qualité générale des emplois vacants et le niveau de qualification et d'expérience des personnes privées d'emploi, le « marché du logement », lui, souffre d'un mal inverse : l'offre est abondante en logements intermédiaires ou à loyer libre, mais la demande se situe plutôt dans les couches sociales les plus modestes, et bien souvent les plus vulnérables.

notamment de l'aide aux maires bâtisseurs ; il semble donc parfaitement inconséquent de chercher à réduire l'importance de ce parc locatif en procédant à des cessions d'immeubles et de biens dont l'existence se révèle pourtant utile au regard des flux de demandes de logement. La vente de logements locatifs n'a sans doute pas à être interdite par principe.

La vente d'un ensemble HLM engendre naturellement la constitution d'une copropriété dont le fonctionnement optimal ne peut résulter que de l'implication consciente et vigilante des anciens locataires devenus accédants à la propriété. Au demeurant, comme le vendeur aura oublié de procéder au reversement des provisions « grosses réparations » d'ores et déjà capitalisées sur l'immeuble, ce sont les accédants propriétaires de leur dette qui se retrouveront le plus souvent avec des choix difficiles d'investissement à financer. Cela n'est qu'un des problèmes qui ne peuvent manquer de se poser dans le cas précis. On notera aussi que l'individualisation des charges locatives de l'immeuble aura, entre autres effets, de majorer sur la durée lesdites charges. Et le processus, quasi inéluctable, de mise en location d'une partie de la copropriété conduira sans doute à de nouvelles difficultés, notamment si les contrats de location sont signés en agence.

c'est-à-dire dire la constitution de copropriétés ingérables ou mal gérées par des syndics vite dépassés par la situation de « propriétaires » endettés pour un logement vite trop petit et parfois aussi rapidement remis en location ou sous-location. Sans compter les externalités négatives nées d'une progression globale des loyers qui a détourné, depuis 1986, une bonne partie de l'épargne des ménages comme des ressources des entreprises du financement de l'économie productive. La parole

à défaut, j'émettrai un avis défavorable. Je ne comprends pas pourquoi on limiterait les compétences des organismes à l'accord du maire. La commission a permis aux organismes d'intervenir plus généralement en matière de revitalisation des centres-villes.

et que son seul recours soit de vendre les logements restants à un organisme d'HLM, associé ou non de ladite société, qui peut dès lors les réintégrer dans le parc locatif social.

pour présenter l'amendement n° 709 rectifié. L'article 28 étend de manière significative les activités que les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent exercer par eux-mêmes ou par le biais de filiales. Or ces nouvelles activités ne relèvent pas du service public d'intérêt général du logement social et sont habituellement exercées par des prestataires de droit privé. La création de ces nouvelles compétences octroyées aux bailleurs sociaux est justifiée par le fait qu'il existerait des zones en carence. Aussi, et c'est l'objet de cet amendement, il convient de préciser dans la loi que ces compétences nouvelles seront limitées aux cas de carence avérée du secteur privé.

chargée de fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Chacun le sait, dans tous nos départements, des services médico-sociaux interviennent déjà régulièrement sur tout le territoire à domicile auprès des personnes en situation de handicap, enfants ou adultes, ou des personnes âgées. Ils assurent aussi des prestations d'accompagnement qui visent notamment à la préservation et la restauration de l'autonomie. En l'état actuel, l'article 28 induit une confusion réelle, en particulier au regard des missions assurées déjà par de nombreux services d'accompagnement à la vie sociale. Il risque par conséquent d'être inopérant, de faire porter aux bailleurs sociaux des missions normalement dévolues à de tels services, qui nécessitent une autorisation spécifique aux termes des dispositions du code de l'action sociale et des familles. Cet amendement vise à interdire une telle ouverture, mais à faire en sorte de ne pas fragmenter l'accompagnement des personnes concernées ; il faut au contraire trouver des synergies avec les services existants. Nous proposons donc de formaliser par convention cette coopération avec l'ensemble des services qui existent déjà sur nos territoires.

L'article 28 comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social. Ainsi, le projet de loi dote les organismes sociaux de nouvelles compétences en prévoyant la possibilité de création de filiales de prestations de services intervenant dans le champ concurrentiel concurrentiel et sans aucune précision concernant les règles et modalités de construction de ces structures. Des filiales pour répondre à des besoins précis, par exemple ingénierie urbaine ou services de gestion, dont la fourniture de services de gestion adaptée aux personnes âgées ou en situation de handicap. handicap. Les filiales créées par les bailleurs sociaux seraient en mesure de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel, réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études d'ingénierie urbaine fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d'un logement social répondant à des besoins « non satisfaits ou partiellement satisfaits On peut s'interroger, d'une part, sur le bien-fondé de cette disposition consacrant les bailleurs dans des missions bien éloignées des leurs et à l'opposé de leurs interpellations sur ce projet de loi part, sur la mise en place de ces services développés sans cahier des charges. Cet amendement vise donc à préciser les modalités d'organisation de ces nouveaux services, en les soumettant à un cahier des charges défini par arrêté ministériel. La fourniture de services à des personnes fragilisées doit être cadrée nationalement, afin de garantir l'égalité de traitement sur tout le territoire.

En plus, je m'interroge véritablement sur les modalités d'application de cette disposition. L'obligation d'avoir une comptabilité séparée entre les activités relevant du SIEG- service d'intérêt

en matière de fourniture de services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou handicapées locataires est réalisé en coordination avec les services d'accompagnement à la vie sociale. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement Enfin, les auteurs de l'amendement n° 173 souhaitent indiquer que l'exercice de la compétence des organismes en matière de fourniture de services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou handicapées locataires est réalisé sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel. Cette activité annexe est soumise à une logique d'offre de service délivrée dans des conditions concurrentielles. Il ne me paraît pas souhaitable

Cet amendement vise à restreindre la possibilité donnée aux organismes d'HLM de fournir des prestations complémentaires en faveur de personnes en perte d'autonomie.

l'accompagnement social des personnes en perte d'autonomie est effectivement un enjeu de société. Les bailleurs sociaux peuvent jouer un rôle important, notamment en direction de leurs propres locataires, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas. Cela peut être un apport précieux sur certains territoires. Toutefois, si ces services entraient dans le champ d'activité soumis à autorisation ou agrément au titre du droit social,

tenons à ce que le travail des bailleurs se fasse en lien avec les collectivités locales. Absolument ! Vous proposez non pas de supprimer cette opportunité, mais d'obliger que cette action se mène au travers d'une convention avec les acteurs, notamment départementaux. Il y a des endroits où c'est utile. En tout état de cause, une telle action doit être coordonnée, que ce soit pour la gérontologie ou pour les personnes en situation de handicap. Nous, nous voterons donc cet amendement.

l'amendement n° 174 rectifié. L'article 28 permet aux offices publics de l'habitat- OPH -, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, de réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière. Ces nouvelles activités ne porteront pas uniquement sur des logements. Cet élargissement du champ de compétences des OPH se fera au détriment de l'ensemble des prestataires de droit privé intervenant dans les mêmes champs d'activité. Cette mesure opérant un transfert de maîtrise d'ouvrage, il convient de préciser que le bailleur social doit, dans ce cadre, respecter les règles de passation et d'exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment celles de la loi MOP qui, sans cela, sera purement et simplement vidée de sa substance. Rappelons que la loi MOP structure les relations entre les acteurs de l'acte de construire, garantit leur indépendance, responsabilise la maîtrise d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre en imposant à ces derniers des obligations de résultat. Dès lors, la remise en cause des règles de la commande publique et de la loi MOP ou la création de nouvelles dérogations ne peuvent que nuire à la qualité

qui pourront, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence messieurs les ministres, cela ne doit pas être un tour de passe-passe. Il ne faut donc pas que les nouvelles activités que pourront exercer les organismes de logement social

OPH pourrait se faire au détriment de l'ensemble des prestataires de droit privé intervenant dans les mêmes champs d'activité. Il nous paraît donc absolument nécessaire de préciser que, dans ce cadre, le bailleur social doit respecter les règles de passation et d'exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment les règles qui régissent la concurrence, le libre accès aux marchés publics et les règles relatives aux concours, en particulier pour l'architecture. En clair, toutes les règles qui sont inscrites dans la loi MOP.

ne puisse pas servir à des dérogations totalement injustifiées au droit commun, qui, en vertu tout particulièrement de la loi MOP, s'applique aux collectivités locales.

Il n'apparaît pas comme possible d'appliquer aux organismes de logement social qui assureront des opérations de construction ou d'aménagement pour le compte de leur collectivité de rattachement les règles applicables à celle-ci, car en droit des marchés publics les règles applicables sont déterminées en fonction de la nature juridique de l'acheteur. Absolument ! Du reste, en tout état de cause, le droit de la commande publique s'applique déjà aux offices publics de l'habitat,

Disons les choses telles qu'elles sont : il faut rassurer. Ces amendements précisent que le bailleur social doit respecter les règles de passation des marchés applicables à la collectivité territoriale de rattachement.

ces offices agiront pour le compte de collectivités locales, pour toute construction susceptible d'être faite dans tout domaine par les collectivités locales, s'appliqueront les règles qui s'appliquent en l'occurrence aux collectivités locales

qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu'au départ des locataires en place. Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu'à l'expiration des baux en place.

Il prévoit en outre d'affecter le surplus des sommes perçues par les organismes vendeurs à des actions et à des opérations de rénovation urbaine.

prenne en compte « les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies Cette disposition a été renforcée par la circulaire du 8 mars 2017 demandant une meilleure prise en compte des femmes victimes de violences dans les obligations imparties sur les logements réservés. Cet amendement vise à renforcer l'action publique en termes d'accompagnement de ces victimes dont la condition socio-économique et le manque d'accès à une aide juridique conditionnent encore trop souvent la décision de quitter une situation conjugale conjugale ou familiale dangereuse. Après l'allocation d'un logement social, les services de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement mentionnés à l'alinéa 29 offriraient un soutien important à des personnes en situation d'extrême fragilité et pour lesquelles tout est à reconstruire.

adoptée à l'Assemblée nationale permettant le rattachement de deux offices publics de l'habitat à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public territorial lorsqu'il existait au préalable sur le territoire plus de cinq offices publics de l'habitat.

est concerné par cette disposition. Rien ne justifie une telle inégalité de traitement, d'autant que les autres dispositions de cet article permettent de conserver le rattachement de plusieurs offices dès lors qu'un seul d'entre eux gère moins de 10 000 logements sociaux, soit le seuil que nous avons fixé. Par souci d'équité,

mais également que ceux qui ont été conclus postérieurement prennent fin au plus tard à la date d'extinction de l'usufruit.

Un amendement du député Teissier a été adopté lors des débats en séance publique permettant aux organismes d'HLM d'acquérir un programme complet de logements sous ce régime. Cette disposition nous semble extrêmement dangereuse puisqu'elle permettrait au fond aux offices de se dédouaner du respect de la loi MOP pour les constructions de logements sociaux et de sortir des règles de la commande publique. En effet, les promoteurs privés ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles et la facilitation de la VEFA conduit à abaisser l'exigence de qualité des logements construits. Nous souhaitons, pour notre part, harmoniser les normes de construction vers le haut plutôt que vers le bas. Cette disposition, fort heureusement, a été supprimée en commission au sénat. Mais nous considérons qu'il demeure nécessaire de légiférer afin d'encadrer le recours aux VEFA. Nous proposons donc de modifier le code de la construction et de l'habitation pour que les opérations réalisées en VEFA soient contenues quantitativement et qu'elles respectent les règles de la commande publique. Actuellement un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte est autorisé à acquérir en VEFA des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. Jusqu'en 2009, les différentes circulaires relatives à la mise en oeuvre de la politique du logement rappelaient systématiquement que la réalisation de logements locatifs sociaux par la procédure de VEFA était autorisée sous certaines conditions, notamment que « la VEFA présente un caractère minoritaire, aussi bien pour l'organisme que pour le promoteur, ou par rapport à l'opération d'ensemble ». Cet amendement traduit cette exigence, qui est aussi une exigence permettant, par la mixité des programmes, la mixité sociale à une échelle très fine. Le recours aux VEFA doit constituer un outil pour développer la mixité des logements et donc des publics, et non pour contourner les règles de commande publique. Quel est l'avis de la commission ? Contrairement

Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote. Je voterai cet amendement, même si je dois féliciter la commission d'avoir rétabli le système existant des VEFA puisqu'on n'élargit pas à la vente en bloc totale des VEFA. Néanmoins, il est aujourd'hui possible de faire des opérations avec 99 % de VEFA.

Cette société n'a en effet pas vocation à gérer du patrimoine, mais à faire du portage en vue de la revente des logements prioritairement. Le portage par les sociétés de vente d'HLM porte néanmoins des enjeux essentiels en termes de sécurisation de l'accession à la propriété et de pérennité du patrimoine. La société de vente a pour mission de revendre les logements à des ménages modestes et doit, à ce titre, mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement ; elle a également des responsabilités liées à la conservation du patrimoine en sa qualité de propriétaire. la CUS, comporte un volet « politique patrimoniale » et un volet « politique d'accession ». À ce titre la société de vente d'HLM doit rester impliquée dans la vie de l'immeuble et de celle des locataires accédants. L'objectif est bien d'assurer l'accession sociale des locataires dans les meilleures conditions possible et d'éviter la dégradation du patrimoine. Notre amendement prévoit ainsi que la société de vente soit signataire de la CUS. Quel est l'avis de la commission ?

On entend ce qui est dit concernant le rôle de la société de portage. Justement, si nous avons la possibilité de travailler sur cette convention pour faire en sorte de mieux huiler le suivi